n° 1679. L'objet de cet amendement est d'élargir la possibilité de transférer la responsabilité d'une maîtrise d'ouvrage concernant des travaux sur le domaine routier ou en vue de la conservation ou de la sécurisation d'une voie. En d'autres termes, il s'agit d'autoriser une collectivité territoriale à transférer à une autre toute la responsabilité des travaux sur le domaine routier, ce que ne permet pas actuellement la rigidité du principe selon lequel le maître d'ouvrage ne peut se départir de sa mission. La pratique a montré que deux types de situations concrètes nécessitent cette souplesse. Dans un premier cas, il peut paraître opportun qu'une collectivité intervienne sur une route appartenant à une autre collectivité, par exemple quand une portion de route ou des ponts sont limitrophes de deux collectivités. En outre, une collectivité, pour son propre développement, peut vouloir améliorer l'aménagement d'une route qui ne relève pas de son domaine routier. Ce peut être le cas pour des routes départementales traversant des agglomérations. Enfin, le transfert de maîtrise d'ouvrage permet l'entraide entre collectivités, par exemple entre une commune et un département. Le second type de situation est celui où des travaux doivent être entrepris pour la sécurisation des voies, par exemple pour éviter des glissements de terrain ou des chutes de pierres. C'est alors une lourde responsabilité que les communes doivent assumer, alors qu'il pourrait être tout à fait légitime que le gestionnaire de voirie prenne les travaux en main. Le transfert de maîtrise d'ouvrage se révélera donc utile pour les collectivités et sans contrainte, puisqu'il reposera sur le volontariat, j'y insiste, des collectivités concernées, qui s'accorderont entre elles, par convention, sur les conditions techniques et financières

des compétences sectorisées du transport et suggère un décloisonnement des compétences, ce qui semble indispensable pour appréhender les grands projets qui feront la mobilité de demain. suggère également la mise en place d'un outil approprié permettant d'associer dans une seule entité publique les différents acteurs pouvant y participer. De telles sociétés de financement peuvent constituer des solutions viables financièrement pour réaliser de grands projets d'infrastructures dans des délais raisonnables. À titre d'exemple, M. Jacquin cite le projet d'autoroute A31 ,

serait source de lourdeurs administratives et de couches de gouvernance supplémentaires, alors que la région constitue déjà l'échelon pertinent pour gérer l'allocation des ressources et garantir l'efficacité attendue d'une approche multimodale. En effet, l'article 32 du projet de loi relatif à la lutte contre le dérèglement climatique, dans la version présentée par le Gouvernement, ouvre déjà aux régions la possibilité d'une ressource complémentaire avec l'écocontribution.

que de l'aménagement de l'A31 , dont le financement, pour la section nord, est envisagé sous forme de concession à péage.

à la demande et scolaires, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés. Elles peuvent également adopter des schémas directeurs d'accessibilité. Toutefois, elles ne peuvent être maîtresses d'ouvrage des travaux de sécurisation, d'aménagement ou de mise en accessibilité des points d'arrêt. Comme l'a précisé le Conseil d'État dans un arrêt du 8 octobre 2012, seule la localisation des points d'arrêt et l'information des usagers relèvent de la compétence des autorités organisatrices de transport que sont devenues nos régions. Cet amendement vise donc à leur permettre d'être maîtresses d'ouvrage dans ce type d'aménagement, puisqu'elles sont les plus à même de gérer leurs circuits, donc les aménagements nécessaires.

et pour les collectivités qui s'engageraient dans cette direction. L'autorité de régulation confirme nos craintes, puisqu'elle souligne le risque d'éclatement de la gestion du réseau ferroviaire. Avec cet article, le Gouvernement agit donc comme si des accords de transfert étaient déjà trouvés avec les régions, ce qui n'est pas le cas. Sur fond d'état dégradé du service, et dans l'espoir de sceller le sort des petites lignes, une mission d'expertise a été confiée au préfet Philizot, dans la foulée du rapport Spinetta, qui en proposait à l'époque l'abandon pur et simple.

Ce projet de loi semble ignorer cet état de fait, tout en le sanctuarisant et en y ajoutant la question très spécifique des gares. Cela revient à transférer sans moyens ce patrimoine dégradé aux collectivités et à leur faire endosser la responsabilité de sa non-remise en état. Il ne s'agit pas d'une bagatelle : selon le rapport Spinetta, quelque 750 millions d'euros seraient annuellement consacrés à l'entretien et à la modernisation des lignes de desserte fine du territoire. Lors de l'audition de Patrick Jeantet par le Conseil d'orientation des infrastructures, en janvier 2019, celui-ci précisait que les besoins d'investissement pour restaurer les performances nominales de ces lignes étaient estimés

quatre prochaines années dans le réseau des lignes de desserte fine du territoire pour le maintenir en capacité de fonctionner, soit un quasi-doublement de l'effort. L'État n'étant pas prêt à assumer ce rôle, il se défausse une nouvelle fois sur les régions, dans un chantage que nous pourrions d'ailleurs qualifier d'odieux. C'est pour nous inacceptable. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Madame la présidente, mes chers collègues, je ne suis pas favorable à la suppression de cet article. D'une part, le transfert des petites lignes ferroviaires aux régions a été permis par l'article 172 de la LOM. Plusieurs régions ont déjà manifesté leur intérêt pour ce transfert et engagé des discussions avec SNCF Réseau. C'est par exemple le cas de la région Occitanie. D'autre part, l'article 172 de la LOM comportait certaines ambiguïtés, notamment s'agissant de la possibilité d'inclure dans le transfert des installations de service. L'article 9 permet de clarifier le champ du transfert et d'approfondir le dispositif introduit par la LOM, en permettant le transfert des lignes d'intérêt local et régional en pleine propriété. Je pense que le transfert aux régions est un moyen

et, le cas échéant, ceux de SNCF Gares & Connexions peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs délégataires lorsqu'est transférée à cette collectivité la propriété ou la gestion de certaines lignes ferroviaires. Il nous a paru opportun de réaffirmer que le maillage ferroviaire, particulièrement en milieu rural, devait être garanti. Cet amendement vise donc à poser comme principe le maintien d'un maillage territorial équilibré dans le déploiement de ce mode de déplacement qui est écoresponsable et qui constitue une solution de rechange aux déplacements automobiles.

manquant de précision. Je pense que cette rédaction poserait des difficultés d'application. Les régions qui reprendront la gestion des petites lignes ferroviaires auront besoin de latitude dans l'exercice de leur mission, et il n'apparaît pas opportun de fixer

M. Didier Marie. Nous considérons qu'il est nécessaire de sécuriser le droit des salariés dans des conditions au moins aussi favorables que celles du code du travail, notamment le droit à mettre fin à leur mise à disposition avant la durée maximale visée par le présent texte consacrant une nouvelle forme de mise à disposition exorbitante du droit commun quant à sa durée, il s'agit de confirmer que cela ne fait pas obstacle aux aux droits garantis par le code du travail. Le consentement du salarié à la mise à disposition est un élément substantiel de ces garanties, qui trouve à s'exercer non seulement avant la mise à disposition, qui doit aussi pouvoir être invoqué à tout moment, y compris après une éventuelle période probatoire, compte tenu de la longue durée de cette mise à disposition. En cas de fin de mise à disposition sur l'initiative du salarié, le contrat de travail se poursuit dans son entreprise d'origine, où il retrouve un emploi identique ou un emploi équivalent.

leur initiative, à la mise à disposition. En effet, la durée de cette convention étant particulièrement longue, il convient de permettre à ces agents, s'ils le souhaitent, de réintégrer la SNCF à tout moment.

pour un temps relativement long, pouvant aller jusqu'à vingt ans. Cela ne doit pas se faire au détriment des droits des salariés. Par cet amendement, auquel a contribué la CFDT Cheminots, nous proposons que le salarié dispose bel et bien du droit de mettre fin à sa mise à disposition, de sa propre initiative,

les amendements identiques n 224 et 1262 n'ont pas le même point d'impact, mais ils ont le même objet. Je proposerai donc un avis commun pour ces trois amendements. Leurs dispositions posent, à mon sens, deux difficultés. prévoir les conditions dans lesquelles un salarié met fin à une mise à disposition ne me semble pas relever du rôle du législateur. Ce serait plutôt du niveau réglementaire, et même contractuel. le décret n° 2020-1820, pris pour l'application de l'article 172 de la LOM, prévoit la possibilité pour un salarié ou pour l'entreprise prêteuse de mettre fin à la mise à disposition. Je le rappelle, en application de ce décret, cette possibilité sera également prévue dans la convention de mise à disposition qui sera conclue par chaque salarié. J'ajoute qu'introduire dans la loi la faculté de mettre fin à la mise à disposition à tout moment interroge au regard du principe de la continuité du service public qui s'applique au transport ferroviaire. D'autre part, s'agissant de l'application aux salariés des droits garantis par l'article L. 8241-2 du code du travail,

s'effectue « dans des conditions prévues par le code du travail. » En pratique, comme dans le droit commun, les deux entreprises et le salarié doivent formaliser dans la convention les conditions dans lesquelles la mise à disposition peut prendre fin.

il est inutile de prévoir explicitement la possibilité de compléter des garanties accordées aux salariés par voie conventionnelle, puisque cela relève totalement du droit commun du code du travail.

un peu. Je prends acte des propos de Mme la ministre, qui nous garantit que le code du travail sera totalement respecté et que, à ce titre, effectivement, les salariés qui seront en disponibilité de longue durée pourront réintégrer leur entreprise. Je rappelle que ces amendements sont issus de discussions que nous avons eues avec les partenaires sociaux. Les syndicats manifestent tout de même leur inquiétude, et je pense qu'il sera utile de les rassurer.

qui, en principe, est garantie dans le cas de prêt de main-d'oeuvre encadré par le code du travail. Il tend à sécuriser, dans tous les cas de figure, la continuité des droits des salariés. Cette mesure est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'une mise à disposition de très longue durée. C'est un élément indispensable de la confiance des salariés dans le dispositif, et il convient donc de s'assurer que cette continuité trouvera également à s'appliquer dans le cas d'une mise à disposition au sein d'une collectivité publique et dans le cas d'une entreprise prestataire dont l'activité principale n'entrerait pas dans le champ de la convention collective ferroviaire et du décret socle sur l'organisation et et le temps de travail. Une telle précision vise à confirmer la solution retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question ambivalente du régime du temps de travail d'un salarié mis à disposition. La haute juridiction a décidé, en l'espèce, qu'un régime de travail en vigueur dans l'entreprise d'accueil, mais interdit par la convention collective dont dépend l'entreprise d'origine, ne pouvait de ce fait être appliqué aux salariés mis à disposition.

repos hebdomadaire, jours fériés, etc. -, et ce pour toute la durée de la mise à disposition. Il s'agit concrètement, avec cet amendement inspiré par une contribution de la CFDT Cheminots, de confirmer dans la loi la solution juridictionnelle retenue en 2011 par la Cour de cassation, qui a décidé que l'entreprise d'accueil ne pouvait appliquer un régime de travail interdit par la convention collective de l'entreprise d'origine. La confiance des salariés dans le dispositif de transfert serait renforcée par l'adoption de ces amendements

le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. » Je rappelle que cet article sera applicable aux salariés mis à disposition, comme le prévoit l'article 9 du présent projet de loi.

continuent d'appartenir à l'entreprise prêteuse. Dans ce cadre, ils continuent de bénéficier du dispositif légal, statutaire et conventionnel applicable dans leur entreprise d'origine. Cela ne peut pas être plus clair.

l'amendement n° 719. Cet amendement vise à promouvoir un compromis social positif, qui encadrera les questions ne pouvant être traitées par l'avenant : modalités d'information préalable des salariés, conditions d'appel au volontariat, suivi des salariés pendant leur mise à disposition, conditions de retour dans l'entreprise d'origine, par exemple. Les mises à disposition et les transferts de personnel à partir du groupe public unifié vont se multiplier dans le cadre de divers marchés portant sur le transport de voyageurs ou sur la gestion de ces petites lignes. Il convient que les partenaires sociaux soient incités à fixer un cadre sécurisant pour les salariés, de sorte que ceux-ci puissent s'engager sereinement dans ces transformations. En l'absence de telles garanties, ces changements pourraient être source de blocage. C'est pourquoi nous souhaitons introduire une disposition supplétive réglementaire en cas de défaut d'accord. je vous remercie,

À mon sens, c'est en ménageant un cadre sécurisant pour les salariés qu'on leur permettra de s'engager sereinement dans ces transformations.

des petites lignes ferroviaires. Le dialogue avec les organisations syndicales sera indispensable pour préparer le transfert de personnel et assurer sa fluidité. Toutefois, je m'interroge sur l'opportunité pour le législateur d'intervenir sur ce sujet. L'organisation de la négociation collective, de même que son contenu, relève de la responsabilité de l'entreprise et de sa vie interne. Par ailleurs, je crains qu'inscrire ce type d'obligation dans la loi n'aille dans le sens d'une rigidification de l'organisation du transfert des petites lignes,

de négociation. On pourrait alors accuser l'État de s'immiscer dans une mission qui n'est pas la sienne. vote. Cette fois, nous maintiendrons notre amendement, considérant qu'il ne s'agit pas de remplacer la négociation entre les parties, tant s'en faut

du 29 décembre 2020. Il est question des lignes séparées du réseau, des lignes d'intérêt local fixées réglementairement et de petites lignes dédiées au transport régional, conformément aux compétences de la collectivité bénéficiaire du transfert. correspondre à l'intention de l'article 172 de la LOM, il est également important de rappeler que ce transfert doit être conditionné au maintien d'une utilisation ferroviaire de l'infrastructure, afin d'éviter tout détournement de procédure pour d'autres besoins.

des lignes séparées du réseau, des lignes d'intérêt local fixées réglementairement et des petites lignes dédiées au transport régional. Par ailleurs, nous entendons rappeler que ce transfert doit être conditionné au maintien d'une utilisation ferroviaire

il faut permettre aux régions de prendre en compte les situations locales. L'objectif de l'article 172 de la LOM est de favoriser la revitalisation des petites lignes et leur pleine intégration aux politiques locales d'aménagement. Les régions, en tant qu'autorités organisatrices de transport, sont compétentes pour organiser les mobilités et les services publics de transport sur leur territoire. Il faut donc leur laisser la souplesse nécessaire pour définir sur chaque territoire l'offre de service qu'elles jugent adaptée en fonction des besoins de la population et de nombreuses autres considérations, notamment économiques. Rappelons que les petites lignes ferroviaires constituent une part très importante du réseau ferré dans certaines régions. Ainsi, en Occitanie, les dessertes fines représentent la moitié du réseau. Le maintien du transport de voyageurs n'est pas forcément pertinent sur toutes les lignes transférées. en imposant un cadre de gestion trop rigide, nous risquerions de décourager les régions de demander le transfert des lignes. Si les régions ne disposent d'aucune latitude quant à l'usage qu'elles feront de ce réseau de petites lignes, elles auront peu d'intérêt à en réclamer la gestion. Par conséquent, l'avis de notre

et à conditionner le transfert de certaines catégories de lignes au maintien de services ferroviaires de transport de voyageurs. Cela conduirait à exclure du champ des lignes transférables des lignes actuellement fermées aux circulations ferroviaires, ainsi que les lignes dites « capillaires fret utilisées uniquement pour le transport de marchandises. Par ailleurs, en imposant le maintien de services de transport ferroviaire de personnes de type ferroviaire lourd, on priverait les régions de la possibilité

l'amendement n° 721. Au-delà des besoins de la politique nationale de transports et de ceux de la défense, il convient de garantir que le transfert de lignes permettra de contribuer à la transition écologique, en améliorant le bilan environnemental de l'exploitation antérieure, ou à tout le moins en ne détériorant cet amendement, nous nous inscrivons dans la nécessité de prendre en compte l'impératif écologique dans tous les actes de la vie publique, notamment en matière de transports, secteur qui contribue particulièrement à l'émission de gaz à effet de serre.

En sauvant les petites lignes, nous allons favoriser le report modal. Deuxièmement, en pratique, je m'interroge sur la possibilité d'apprécier l'impact environnemental de chaque transfert. Au moment de demander le transfert de propriété, les régions n'auront pas nécessairement un projet détaillé pour l'avenir de ces lignes. Rappelons également

Néanmoins, adopter ces amendements imposerait d'analyser l'impact d'un projet de transport ferroviaire préalablement au transfert de gestion de la petite ligne en question, ce qui alourdirait les procédures de transfert, alors même que la collectivité intéressée pourrait porter un projet alternatif, mieux adapté aux besoins des territoires desservis, tel que des bus à haut niveau de service en site propre, ou encore des véhicules du type « train très léger ». Il semble donc préférable de ne pas réduire le champ des possibilités offertes aux bénéficiaires des transferts.

dite loi ORTF, a fixé des échéances spécifiques pour l'ouverture à la concurrence des services réguliers de transport guidé en région Île-de-France, ainsi que des services réguliers de transport routier, de transport par tramway et de transport scolaire.

Quant aux lignes de RER A et B gérées par Île-de-France Mobilités, qui sont les services les plus empruntés du réseau, leur ouverture à la concurrence devait avoir lieu en 2039, soit au même moment que pour les services exploités par la RATP. Le présent amendement vise à avancer de dix ans pour la fixer en 2029. Je suis sensible aux arguments selon lesquels une diversification des opérateurs dès 2030 permettra à Île-de-France Mobilités de sélectionner des offres plus adaptées aux besoins et de favoriser une qualité de service optimale pour les usagers. Par ailleurs, l'avancement de ces dates correspond à une demande d'Île-de-France Mobilités. Mme Valérie Pécresse n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler lorsqu'elle a été entendue par notre commission au mois de février dernier. Toutefois, je souhaite émettre une réserve : les délais d'examen du texte qui sont les nôtres ne m'ont pas permis d'entendre les parties prenantes, notamment les opérateurs, ni d'évaluer pleinement les répercussions de cette proposition. Le processus d'ouverture à la concurrence est déjà lancé sur de nombreuses lignes ; modifier le calendrier en cours de route risque donc de déstabiliser les travaux qui ont été lancés.

de l'aménagement du territoire ? L'ouverture à la concurrence des lignes de TER permet aux régions d'avoir recours aux services de la SNCF, opérateur historique, ou de prestataires privés pour la réalisation des services de transport de voyageurs. Dans ce cadre, il est prévu qu'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs soit conclu entre l'autorité organisatrice de transport et l'attributaire. En cas de changement d'attributaire, l'article L. 2121-20 du code des transports prévoit le transfert des contrats de travail en cours depuis au moins six six mois à la date de notification de l'attribution. L'article L. 2121-22 précise les modalités de détermination des effectifs transférables

des salariés concourant directement ou indirectement à l'exploitation du service concerné ». Or les procédures de changement d'attributaire sont souvent longues. Entre le moment salariés à transférer est arrêté et le changement d'attributaire, les effectifs employés peuvent évoluer substantiellement. Cet amendement, qui vise à prendre en compte non pas une photographie des effectifs, mais leur trajectoire prévisionnelle, me semble donc pertinent. Toutefois, compte tenu des effectifs importants

Cet amendement vise à prendre en compte les évolutions prévisibles de l'organisation de la SNCF dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. Il convient cependant de tenir compte, d'une part, de la nécessité de préserver l'égalité de traitement des candidats au regard des règles de la commande publique, et, d'autre part, des conséquences économiques et sociales du calcul de ce nombre d'emplois, qui se révèle déterminant pour les entreprises comme pour les salariés au moment du changement effectif d'attributaire. À ce titre,

Par ailleurs, il me paraît nécessaire d'encadrer davantage les modalités selon lesquelles le nombre d'emplois transférés pourrait tenir compte des évolutions prévisibles de l'organisation de la SNCF, de manière à refléter au mieux le nombre de salariés concernés au moment du transfert. particulier, ces évolutions, quoique prévisionnelles, doivent être suffisamment certaines pour ne pas créer un nouveau décalage entre le nombre d'emplois fixé en amont et le nombre effectif des salariés qui seront transférés au moment du changement effectif d'attributaire.

Aujourd'hui, la situation de ces lignes reste extrêmement précaire, comme le souligne le rapport Philizot. Les lignes de desserte fine du territoire, souvent appelées « petites lignes »,

Notre amendement vise à inclure dans les objectifs de la stratégie et de la programmation financière opérationnelle des investissements de l'État dans les systèmes de transport le renforcement

dont 6,4 milliards d'euros restent à engager à partir de 2020. Les régions ne peuvent engager ces investissements. Nous pensons qu'il est de la responsabilité de l'État de permettre la poursuite de ces lignes de vie pour nos concitoyens, y compris au moyen des contrats de plan. Nous considérons, par conséquent, que l'État doit apporter des réponses financières pertinentes aux collectivités territoriales

Les besoins de financement auxquels feront face les régions seront donc, en principe, couverts. Il n'est pas cohérent de maintenir ce système de financement partagé alors que les lignes reviendront entièrement aux régions. l'objectif qui sous-tend cet amendement est celui du maintien de l'ensemble des petites lignes ferroviaires UIC 7 à 9, qui sont les moins fréquentées du réseau. Or les régions ne souhaiteront peut-être pas maintenir l'ensemble de ces lignes. Il faut leur laisser l'autonomie nécessaire pour décider de leur sort. Prévoir un subventionnement de SNCF Réseau pourrait induire une pression sur les régions en faveur du maintien des lignes. Cela n'est pas cohérent avec l'esprit du transfert.

est à Mme la ministre. L'article 4 de la loi d'orientation des mobilités prévoit la possibilité de créer des établissements publics locaux ayant pour mission de financer, sur un périmètre géographique déterminé, un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant 1 milliard d'euros hors taxes. Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place des services complémentaires ou connexes à celles-ci. Cette disposition a été adoptée pour faciliter l'association des collectivités concernées par les projets à leur conception et à leur financement.

Cela pourrait, par exemple, concerner le projet de ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, prévu en quatre phases et dont le Gouvernement a annoncé le financement au titre des deux premières phases voilà quelques semaines. pour objet d'élargir la possibilité de créer de tels établissements publics locaux pour les projets ayant fait l'objet d'une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l'ouverture de l'enquête publique. Or la loi d'orientation des mobilités ne réserve cette possibilité qu'aux projets ayant ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une déclaration de projet ou d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique et d'une contre-expertise à l'évaluation socioéconomique.

Nous avions adopté ce dispositif dans le cadre de la LOM. Il s'agit ici de l'approfondir pour prendre en compte le cas des grands projets phasés, dont fait effectivement partie la ligne ferroviaire nouvelle Provence-Côte d'Azur, prévue en quatre phases, qui vise à désaturer les noeuds ferroviaires de Marseille, Toulon et Nice et à améliorer les liaisons ferroviaires entre ces métropoles pour faciliter les déplacements quotidiens. Cette proposition va dans le sens du renforcement des moyens à disposition des collectivités territoriales pour mettre en oeuvre et financer les grands projets d'infrastructures.

en réutilisant et réaménageant des lignes de chemin de fer fermées, avec pour objectif la recherche de la baisse des coûts énergétiques, financiers et environnementaux, tout en améliorant la qualité de service aux usagers, pour concurrencer efficacement efficacement l'usage de la voiture. Mon collègue Olivier Jacquin s'appuie sur l'exemple de la région Grand Est, qui soutient, depuis 2017, un projet innovant de transport autonome sur rail. a été développé par les universités et les laboratoires de recherche et conduit aujourd'hui à un nouveau paradigme de déplacement, fondé sur une flottille de petits véhicules autonomes sur rail hyperlégers, pour une ou deux personnes, une personne à mobilité réduite ou une personne et son vélo, qui concurrencent efficacement l'usage de la voiture individuelle.

de complémentarité avec les autres moyens de transport et même d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette solution innovante me semble aussi intéressante au regard d'objectifs de désenclavement et de mise en valeur des zones rurales. Je suis tout à fait favorable au fait de laisser aux régions qui le souhaitent la possibilité d'expérimenter ce type de projets. Cependant, j'ai quelques réserves sur le délai de deux ans qui est proposé : puisque les lignes ferroviaires concernées nécessiteront d'importants travaux, cette durée me semble courte pour conduire des investissements et permettre la mise en service de ce mode de transport. Par ailleurs, hormis la région Grand Est, qui porte ce projet de transport autonome depuis 2017, je n'ai pas connaissance, à ce stade, de régions intéressées. Je m'en remets donc à la sagesse

vient de livrer son analyse de la politique de sécurité routière. Elle critique notamment la politique répressive du tout-radar, qui ne permettrait pas de limiter le nombre d'accidents chaque année, constatant même un essoufflement de ces méthodes. La Cour encourage la sécurisation des infrastructures, au lieu de se focaliser sur le comportement des individus. À contre-courant de ce rapport, l'article 10 du projet de loi, dont nous proposons la suppression, permet aux collectivités d'installer des radars automatiques.

être étudiée dans le contexte actuel. À la critique de l'efficacité des appareils s'ajoute une baisse du produit des amendes d'au moins 12 % en 2019, ainsi qu'une hausse des coûts d'investissement pour remplacer les appareils endommagés et en déployer de nouveaux. Les collectivités pourraient se retrouver face à un réel risque financier avec cette nouvelle compétence, devant assumer de nouvelles charges d'installation et d'entretien. Rappelons également que le produit des amendes n'est que partiellement reversé aux collectivités et que, en l'état, nous ne disposons pas d'informations détaillées sur le bénéfice d'un tel transfert pour les collectivités, d'autant plus qu'aucune subvention ne semble prévue pour ces financements nouveaux.

Ensuite, la disposition soulève des difficultés pratiques, auxquelles le Gouvernement n'apporte pas de réponse, puisque tout est renvoyé à un décret en Conseil d'État. L'article qui ouvre cette faculté à toutes les collectivités et à l'ensemble de leurs groupements ne prévoit notamment pas de mécanisme destiné à assurer la cohérence de l'implantation des radars. On pourrait imaginer qu'un conducteur sortant du périmètre d'une commune et entrant dans une autre

que le traitement des constatations effectuées par ces appareils répond à des modalités identiques à celles qu'effectuent les radars installés par l'État.

qui étend ses dispositions aux collectivités d'outre-mer du Pacifique. En effet, le dispositif national de contrôle automatisé des infractions détectées par les radars n'y est pas installé. L'amendement n°

! L'article 10 prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à installer des appareils de contrôle automatique. En revanche, il ne prévoit pas qu'ils soient intéressés aux recettes issues des amendes, alors même que l'installation de ces équipements représente une charge financière considérable pour les communes. Aussi, il semble opportun que les modalités de répartition des recettes tirées de ces contrôles soient définies par décret en Conseil d'État, afin de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier de tout ou partie des recettes issues des appareils de contrôle installés à leurs frais sur leur territoire. Quel

Or il est actuellement impossible de vérifier de manière objective que l'usager paie effectivement le tarif correspondant à l'impact réel de son véhicule sur la pollution atmosphérique, et la multiplication des contrôles visuels par des agents sur le terrain représente une charge trop importante pour les collectivités. Afin que les collectivités puissent disposer des informations indispensables à l'application d'une tarification adaptée aux véhicules, les maires doivent pouvoir recourir au fichier national du système d'immatriculation des véhicules. Cet accès permettrait entre autres

abordé la question des conflits de légitimité entre la métropole de Lyon et un certain nombre de communes, du fait d'une élection au scrutin direct pour la métropole et d'un scrutin identique pour les communes. Le sujet du stationnement est récurrent. En effet, un certain nombre

qu'à partir du moment où il existe une délibération concordante du conseil municipal.

En l'état actuel du droit, les appareils photographiques mobiles ou fixes prenant uniquement des photos par déclenchement automatique lors de la détection d'un passage par la cellule de l'appareil n'entrent pas dans le champ d'application de la réglementation des dispositifs de vidéoprotection. Afin de permettre la constatation d'infractions, notamment environnementales- dépôts sauvages en milieu naturel, vols sur les exploitations agricoles, et j'en passe -, qui empoisonnent la vie des citoyens et des maires, il est important d'outiller les gardes champêtres d'appareils photographiques, de manière à établir la réalité de l'infraction. Pour garantir le droit au respect de la vie privée, la mise en place de tels dispositifs sera soumise à l'autorisation du ou des propriétaires des terrains concernés et à l'information préalable du procureur de la République, qui pourra s'y opposer. Enfin, les prises de vues obtenues n'auront d'autre but que d'appuyer les constats opérés, ne recevront aucune utilisation publique et seront couvertes par le secret

dans la mesure où le dispositif limite l'usage de tels dispositifs à une catégorie d'agents pour des infractions délimitées et dans des lieux restreints, dont la définition ne paraît pas très précise, il pourrait en résulter une interdiction de certains usages aujourd'hui possibles dans d'autres situations. Par ailleurs, si l'utilisation de ces dispositifs ne relève pas du cadre juridique de la vidéoprotection, il ne paraît pas nécessaire de prévoir un encadrement juridique spécifique, dans la mesure où, en matière pénale et sauf loi contraire, l'administration de la preuve est libre. Dès lors, tout élément de preuve résultant de l'usage, dans des conditions loyales, d'un appareil photographique fixe ou mobile par les gardes champêtres est recevable par la juridiction compétente.

Une mission de préfiguration de la création d'un établissement public portuaire à Saint-Pierre-et-Miquelon commencera le 1juillet 2021, pour une durée de six mois. Cette mission examinera les modalités d'association de la collectivité à la gestion du port.

Or ces acteurs locaux sont des intervenants essentiels, notamment dans le secteur rural, et ils participent déjà activement à la conduite des politiques publiques en matière de transition écologique : je pense aux acteurs des projets alimentaires territoriaux et de la rénovation énergétique

étroit avec les politiques menées par les collectivités et les projets qu'elles développent. Nos collectivités locales, en particulier nos communes, sont en effet de plus en plus engagées dans la transition écologique. Il convient qu'elles soient représentées dans toute leur diversité au sein de l'Ademe. l'Ademe. Cet amendement tend donc à ajouter, aux côtés des actuels représentants désignés, un représentant des communes de 10 000 à 100 000 habitants, lesquelles sont très actives dans les politiques de transition écologique,

une représentation équilibrée des différentes parties prenantes. Si l'article 12 de la loi tend à ouvrir le conseil d'administration aux EPCI, l'étude d'impact prévoit que « le nombre de représentants pour ce collège resterait de trois ce qui rend cette ouverture quasi inopérante. Cet amendement vise donc à permettre réellement la représentation des différents échelons des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui sont fortement impliqués dans les politiques de transition écologique, et des partenaires de l'Ademe, cela sans exclusive de leurs caractéristiques. Il est difficile d'imaginer que les mêmes administrateurs puissent représenter de manière pertinente les métropoles, les communautés de communes en milieu rural

En revanche, je vous indique que le Gouvernement réservera un siège supplémentaire aux intercommunalités par voie réglementaire. Cela portera la représentation des collectivités à 16 %, ce taux étant assez

Un tel dispositif, qui permet aux régions de disposer de l'ensemble des fonds précités, et non simplement d'un cinquième de leurs montants comme le prévoyait le texte initial, nous semble remettre en cause la cohérence de l'action de l'Ademe à l'échelon national, notamment en termes de pilotage. En effet, une fois qu'elle

régions. La concertation que j'ai menée dans tous les territoires pour préparer le présent projet de loi a fait émerger le besoin de renforcer les compétences et les moyens d'action des régions en matière d'économie circulaire et d'énergies renouvelables. En effet, les régions disposent de moyens limités dans ces domaines, alors qu'elles sont chefs de file en matière d'énergie et de climat. Elles jouent un rôle important dans le financement des projets

L'Ademe, en sa qualité d'établissement public autonome, doit conserver un pouvoir d'appréciation et de décision s'agissant de compétences qui lui ont été confiées par le législateur. L'objet du présent amendement est de rétablir une rédaction plus appropriée et plus respectueuse de l'autonomie de l'Ademe.

la conclusion d'une convention qui fixe, entre autres, les objectifs à atteindre. Cet amendement tend à prévoir que la région associe les autres collectivités, qui participent également à ces politiques vertueuses et connaissent les spécificités locales, ainsi que les besoins des territoires, à l'instruction et à l'octroi des aides et des concours financiers.

notamment l'habitat. Elles sont réparties sur l'ensemble du territoire national et contribuent à déployer des actions de conseil et d'assistance pour réduire les consommations et dépenses d'énergie, favoriser la production d'énergies renouvelables, lutter contre la précarisation des habitats les émissions de gaz à effet de serre. Les ALEC sont actuellement sous pression, comme l'a récemment rappelé Emmanuelle Wargon. En cette période de forte demande de rénovation énergétique, la question de leur capacité à accompagner les ménages est en effet essentielle.

Cet amendement du président Requier vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l'énergie et du climat et à répondre aux besoins de proximité et d'efficacité attendue par les élus locaux. Ces agences constituent un modèle particulièrement pertinent pour accélérer la transition énergétique des territoires. Créées et animées par les collectivités territoriales, elles accompagnent quotidiennement les territoires pour une meilleure prise en compte des questions d'énergie et de climat dans leurs champs de compétences, tant sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel, notamment grâce à l'ingénierie territoriale qu'elles proposent aux particuliers et aux collectivités. L'adoption de cet amendement permettrait de renforcer les outils à disposition des élus locaux pour accélérer la transition écologique dans leurs territoires.

Présidées par le préfet du département, elles regroupent, outre des élus, des représentants de l'État, des professions agricoles et forestières, des chambres d'agriculture, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers et des associations. Cette

Renforcer le poids des collectivités territoriales en attribuant au moins 50 % des sièges à leurs représentants, comme le prévoit l'article 12 , reviendrait mathématiquement à amoindrir la représentation des autres acteurs, qui pourraient

Ces commissions n'entravent pas les élus dans leur prise de décisions, puisqu'elles émettent essentiellement des avis simples, faiblement contraignants, les avis conformes concernant essentiellement les atteintes substantielles aux productions sous appellation d'origine protégée.

madame la ministre,

pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 ne permet pas aux CDPENAF d'être consultées, même de manière facultative, sur les plans locaux d'urbanisme (PLU), dès lors que les communes concernées sont situées dans le périmètre d'un schéma

Les schémas adoptés après 2014 sont ainsi globalement vertueux en matière de consommation d'espace. Néanmoins, c'est au niveau du PLU que s'apprécient finement les différentes implications relatives à la consommation d'espace. Il existe en effet une différence d'échelle, de précision et d'opposabilité entre un SCoT, qui porte sur un large territoire, et un PLU, qui s'attache à l'échelle cadastrale. À cette échelle, la CDPENAF peut s'assurer que la collectivité a bien mobilisé l'ensemble des solutions visant à minimiser la consommation et à maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers. La mesure proposée est ciblée

prévoit qu'un règlement intérieur, dont le contenu serait fixé par décret, assure, entre autres choses, une information suffisante des membres de la commission sur leurs droits, leurs obligations et les avis qu'ils

pas seulement pour les sites exclusivement terrestres. L'ajout de cette consultation a un sens s'agissant des sites exclusivement terrestres, dont la gestion est décentralisée à l'échelon régional, mais cette consultation supplémentaire n'est pas opportune autres sites, mixtes et marins, qui sont exclus du périmètre de la décentralisation en raison de la compétence exclusive de l'État sur le domaine public maritime. Par conséquent, cette rédaction va à l'encontre du principe de simplification que nous défendons dans ce projet de loi. outre, les alinéas 4 et 5 de l'article 13 attribuent au conseil régional la possibilité de proposer, après consultation des communes et EPCI, la création ou la modification de périmètre d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre. Le conseil régional, au même titre que toute collectivité territoriale, peut déjà soumettre un projet de création ou de modification d'un site Natura 2000. De surcroît, la procédure de création ou de modification d'un site Natura 2000 comporte déjà une phase de consultation des communes et des EPCI. Cette redondance ne nous semble pas utile.

d'un site Natura 2000. L'alinéa 3 de l'article 13 prévoit que, dans le cadre de la procédure de délimitation du périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du conseil régional sera désormais demandé au même titre que celui des organes délibérants des communes et des EPCI concernés, comme le prévoit actuellement le III de l'article L. 414-1 du code de l'environnement. Les sénateurs du groupe socialiste estiment nécessaire d'associer également les conseils départementaux dont les territoires sont concernés par la création d'un site Natura 2000- ils sont aujourd'hui occultés de cette procédure de consultation.

En effet, il revient sur la position adoptée en commission qui permet aux conseils régionaux d'être forces de proposition en matière de création de sites. En ce qui concerne les redondances dans la procédure de consultation, les projets soumis par l'autorité compétente de l'État aux collectivités territoriales ne seront pas nécessairement identiques à ceux qui sont proposés par le conseil régional. Il pourra donc être pertinent de consulter les collectivités avant la notification de la proposition à la Commission européenne. nous pourrions clarifier la rédaction, en prévoyant que, lorsque le préfet soumet à la Commission européenne le projet proposé par la région, la consultation n'est pas nécessaire- nous pourrions y retravailler dans le cadre de la navette. L'amendement n° 541 L'amendement n° 541 vise à ouvrir la consultation préalable à la création d'un site Natura 2000 aux départements. Celle-ci est déjà ouverte aux communes et groupements concernés et le projet de loi prévoit de l'étendre aux conseils régionaux. Il paraît logique d'inclure le département dans cette phase consultative, d'autant plus que les départements exercent également des compétences en matière de protection de l'environnement. Ils sont d'ailleurs compétents pour mettre en oeuvre la politique des espaces naturels sensibles, lesquels peuvent parfois se situer sur des sites Natura 2000. Il me semble dès lors légitime que les départements soient consultés dans la phase de création de sites Natura 2000. L'avis est donc favorable

Natura 2000. Cette fois, il s'agit de prévoir la consultation du conseil départemental préalablement à la présentation par le conseil régional d'un projet de création de site à l'autorité compétente de l'État.

C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à ce que les régions soient

des gestionnaires d'aires protégées dans les comités de pilotage des sites Natura 2000. Il s'agit d'instaurer davantage de dialogue entre les réseaux d'aires protégées afin que les différents enjeux écologiques et sociétaux écologiques et sociétaux soient mieux pris en compte. Cet amendement ouvre également la possibilité de confier la responsabilité de l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre à une structure gestionnaire,

Il est important que les régions, qui deviendront autorité compétente à partir du 1 janvier 2023 à la place des préfets de département, puissent bénéficier de l'expertise et du soutien des structures gestionnaires ayant une expérience confirmée dans l'animation de sites

les gestionnaires des espaces naturels protégés dans les comités de pilotage Natura 2000, lorsqu'un site couvre d'autres espaces protégés.

Il s'agit, dans un souci d'efficacité, de les associer étroitement à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre des documents d'objectifs qui déterminent les mesures spécifiques de prévention, de conservation et de rétablissement des habitats et des populations, dont les sites Natura 2000 font l'objet.

à une structure gestionnaire, lorsqu'aucune collectivité territoriale ou aucun groupement de collectivités territoriales ne souhaite être la structure porteuse et que cette fonction est, de ce fait, assumée par l'autorité administrative. Il permet de garantir l'élaboration de documents d'objectifs et leur animation par des structures gestionnaires compétentes ayant les capacités pour assumer des missions très diversifiées. Son objectif est également de renforcer l'action publique en matière de biodiversité grâce à une meilleure prise en compte des enjeux écologiques et sociétaux présents dans les sites Natura 2000.

les gestionnaires des aires protégées au comité de pilotage Natura 2000, lorsque le site couvre d'autres espaces protégés. Ils visent également à confier à une structure gestionnaire la possibilité d'élaborer et d'animer la mise en oeuvre du document d'objectifs qui définit les mesures et orientations relatives à la gestion Sous couvert d'un souci de bonne administration, cette disposition risque selon moi de diluer le rôle des collectivités au sein du comité de pilotage et de le déséquilibrer en faveur des associations agréées qui sont parfois gestionnaires d'espaces naturels protégés. Par ailleurs, je crains que l'intégration de ces représentants au sein du comité de pilotage ne ralentisse la prise de décision et ne complexifie les procédures. Je n'y suis donc pas favorable. En conséquence, je ne suis pas non plus favorable à l'idée d'habiliter ces structures à élaborer et animer la mise en oeuvre du document d'objectifs. Cela reviendrait à dessaisir la région

droit en vigueur. Ainsi, la participation des gestionnaires des espaces naturels protégés est prévue par les textes, en application de l'article R. 414-8 du code de l'environnement. Cet article précise que le comité de pilotage comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants d'organismes exerçant leur activité dans le domaine de la prévention du patrimoine naturel.

Ensuite, si l'autorité administrative qui pilote le site Natura 2000 souhaite déléguer la rédaction du document d'objectifs, elle engage une procédure de marché public à laquelle les gestionnaires d'espaces protégés peuvent répondre- c'est une pratique courante. Au nom du respect des principes de la commande publique- transparence, égalité de traitement et liberté d'accès -, il n'est pas envisageable de dispenser les gestionnaires d'espaces protégés de cette formalité de procédure.

Le code général des collectivités territoriales impose aux collectivités territoriales une participation minimale au financement des projets d'investissement dont elles sont maîtres d'ouvrage. Cette participation est fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques au projet. Or cette obligation d'autofinancement est un frein à la signature des contrats Natura 2000 et plus généralement aux opérations en faveur de la biodiversité menées en déclinaison des documents de gestion de ces aires protégées. Par exemple, les très petites communes n'ont pas les moyens financiers suffisants pour assurer le financement minimal de ces travaux. Malgré les nombreux cofinanceurs prêts à aider les communes, il a été constaté, à de nombreuses reprises, que cette disposition était un frein à l'exécution de ces travaux. Il est donc proposé, par cet amendement, de permettre au préfet de département d'accorder une dérogation à l'obligation d'autofinancement pour la réalisation de travaux répondant à un objectif de préservation ou de restauration de la biodiversité et effectués dans une aire protégée. Je vous remercie,

Le présent amendement vise à supprimer l'article 13 adopté par la commission des lois du Sénat. Cet article introduit une dérogation à la règle de participation minimale du maître d'ouvrage au financement d'une opération d'investissement, en permettant au préfet de département ou au président du conseil régional de réduire le taux de participation minimale de 20 % des communes ou de leurs groupements,

Enfin, une telle dérogation serait déresponsabilisante pour les collectivités qui doivent nécessairement avoir les moyens de financer en partie leurs investissements. Il s'agit d'une règle saine de gestion publique.

Au niveau national, les financements de l'Office français de la biodiversité comme ceux des agences de l'eau peuvent, de la même manière, soutenir les projets des collectivités. Enfin, le Gouvernement a récemment créé une dotation de soutien à la protection de la biodiversité

Cet amendement tend à supprimer l'article 13 portant augmentation de la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés dans un site Natura 2000 faisant l'objet d'un engagement de gestion. Cette disposition relève du domaine de la loi de finances, puisqu'elle augmente les compensations d'exonérations versées par l'État aux collectivités. En outre, elle nécessite une évaluation préalable de son coût.

Les dispositions du plan Loup, que nous approuvons, permettent, à titre dérogatoire et sous le contrôle de la Commission européenne, de réguler sa présence des autorisations de prélèvement délivrées par le préfet.

Toute dérogation supplémentaire doit faire l'objet d'une justification auprès de la Commission européenne. Il est du reste fort peu probable que le présent article soit en conformité avec le droit européen.

Si la régulation est nécessaire, elle ne peut s'envisager qu'à l'échelon national. Le présent dispositif semble parfaitement inopérant de ce point

Le nombre de loups est loin d'être stabilisé en France : il ne convient pas pour l'heure de prévoir d'autres dérogations au plan Loup.

et de l'État, sur la politique spécifique à conduire en faveur du développement durable des massifs. Pour le dire autrement, ils exercent la fonction de conseil économique et social de la montagne. Aussi, nous croyons que les attributions de cette instance de concertation doivent être renforcées. Dans cette perspective, l'amendement déposé sur l'initiative de mon collègue Jean-Yves Roux vise à prendre en compte l'avis du comité de massif concerné avant la publication d'un arrêté motivé par le préfet, dès lors que la réglementation ou l'interdiction d'accès à des espaces naturels protégés concerne plusieurs communes de montagne du massif.

pour s'adapter aux situations locales. Je suis certaine que les gestionnaires d'espaces protégés, qui seront associés naturellement à ce nouveau dispositif, ne seront pas gênés dans leur mission. Je mets aux voix

ou du président de l'EPCI compétent en matière d'environnement et de lutte contre les nuisances sonores sur son territoire. Il ambitionne de renforcer l'action publique locale, en proposant une solution à la disposition des communes et des EPCI compétents en matière d'urbanisme, afin de lutter contre les nuisances, notamment environnementales, qui sont liées à l'usage banalisé de l'hélicoptère.

concerné puisse réguler le trafic d'hélicoptères sur son territoire. Cet outil de planification contribue aux objectifs de préservation de l'environnement, au sens de l'article L. 571-7 du code de l'environnement, en vertu du principe

Quel est l'avis du Gouvernement ? Je ne suis pas non plus une experte en hélicoptères. La réglementation actuelle, à travers les documents de planification existants, permet déjà de concilier le trafic des hélicoptères et certaines préoccupations, que l'on comprend parfaitement, relatives à la sécurité, la sûreté et l'environnement. L'attribution d'une telle compétence à l'échelon intercommunal ne me paraît pas adaptée, car les enjeux liés au trafic d'hélicoptères dépassent bien souvent ce périmètre intercommunal.

Mme Dominique Vérien. À l'été 2020, les espaces nationaux protégés ont été plébiscités par les touristes français. De nombreux sites naturels protégés ont ainsi été confrontés à une hausse inédite des visiteurs pendant plusieurs semaines,

par la réglementation sur les sites classés. Dans l'urgence, il leur a été impossible de réaliser de tels projets, comme des aires de stationnement, puisque la réalisation d'aménagements temporaires ne peut excéder quinze jours, selon les dispositions réglementaires prévues dans le code de l'urbanisme. Pire, cette rigidité risque de conduire à des aménagements temporaires de qualité médiocre. Le présent amendement vise à élargir le champ de la dispense de toute formalité aux constructions, aménagements, installations et travaux réalisés

protégés. Les aménagements temporaires envisagés dans le dispositif de l'amendement sont déjà rendus possibles par le code de l'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire de le modifier. Leur durée est effectivement limitée à quinze jours. L'évolution de ce délai

elles n'ont pas vocation à perdurer trop longtemps. Dispenser de formalités les travaux pérennes réalisés sur ces sites serait totalement contraire à l'objectif de préservation des espaces naturels, plus particulièrement en secteur protégé,

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que, « lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. Mes chers